mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le 13 mai dernier, nous apprenions avec une profonde tristesse le décès de notre ancien collègue Jean Faure. Profondément enraciné dans son Vercors qu'il aimait tant, il fut maire d'Autrans pendant un quart de siècle, vice-président du conseil général, conseiller régional et, en 1983, il fut élu sénateur de l'Isère, mandat qu'il exerça avec exemplarité et conviction jusqu'en 2011. Pour lui, notre assemblée était- je le cite -« une école de la vie ». Il fut un grand sénateur. En témoigne l'affection que tous ses collègues, quelle que soit leur appartenance politique, lui portaient. Il siégea à son arrivée au sein du groupe de l'Union centriste des démocrates de progrès, puis au groupe de l'Union Centriste et, enfin, au groupe UMP. En témoignent également les éminentes fonctions qui lui furent confiées au Sénat : secrétaire du bureau, vice-président du Sénat, questeur. Il présida à lui seul plus de 2 000 heures de séance. En témoignent En témoignent enfin ses combats, tout d'abord au sein de la commission des affaires économiques, puis au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Toute sa vie, Jean Faure puisa dans cette sagesse son humanisme, dont nous garderons le souvenir. J'ai eu l'occasion de lui rendre hommage le 18 mai dernier à Autrans, au milieu de ses montagnes, en présence de ses proches, des élus et de sa famille. Je voudrais associer au moment de recueillement que nous allons observer trois autres anciens collègues qui, malheureusement, nous ont quittés depuis la suspension de nos travaux en mars

Dans la tradition du Sénat, et au nom du bureau, j'appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles pour nous au Sénat : le respect.

Cette situation était pourtant prévisible. En février, nous vous alertions sur le probable blackout et nous avions formulé douze recommandations. Pas de réponse, évidemment. Surtout, nous avons perdu dix ans : dix ans d'une politique énergétique qui s'est acharnée, comme nous l'avons entendu ce matin, à détruire le monde d'hier

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la présidente Primas, nous sommes aujourd'hui confrontés à l'une des pires crises énergétiques depuis le choc pétrolier des années 1970.

construire l'électricité et le monde décarboné de demain : la canicule nous rappelle à quel point il est urgent de s'y investir. Nous agissons, d'abord en mobilisant tous les moyens

leur domaine, les administrations, pour faire cette économie de 10 % qui est absolument nécessaire pour nous décarboner et nous passer des énergies fossiles, et qui nous permettra de passer plus facilement ces moments de crise énergétique.

pour la réplique. Nous voudrions vous croire, mais cela fait dix ans que le Sénat lutte contre des trajectoires qui sont de fausses trajectoires, puisque nous n'atteignons jamais l'objectif. La fermeture de Fessenheim, la réouverture des centrales à charbon sont des exemples de ce manque d'anticipation et de cette fausse route sur l'énergie. Nous voulons des énergies renouvelables, nous voulons des énergies décarbonées, nous voulons la sobriété, mais maintenant, nous voulons des actes

les élus locaux sont accoutumés aux crises de migraine provoquées par la complexité des sujets qui font leur quotidien. Toutefois, l'art de la complexité a atteint un sommet avec la mise en oeuvre du zéro artificialisation nette La sobriété foncière est une nécessité que personne ne discute. Justement, parce qu'elle s'impose à nous tous, il faut s'assurer d'atteindre l'objectif. Or, monsieur le ministre, en l'absence de définition de la chose

accepterez-vous la proposition du Sénat de réviser les conditions de mise en oeuvre du ZAN ? Après l'hommage de Mme la Première ministre à la sagesse inspirante du Sénat, une réponse elle aussi empreinte de sobriété- comme la consommation foncière -sous la forme d'un « oui » serait un très bon début ! La parole est

un risque de disparités dans l'application territoriale. Aujourd'hui, beaucoup d'élus

de la manière dont nous fabriquons la loi. Aucun texte ne devrait être présenté au Parlement sans une étude d'impact complète et systémique, pour que la cohérence des politiques du Gouvernement soit respectée.

Tout cela dépasse le cadre normal des relations entre la puissance publique et les intérêts particuliers de cette entreprise. Si un ministre de l'économie rencontre et échange avec les représentants d'intérêts privés, il n'en oublie jamais le sens de l'intérêt général. Après la privatisation des décisions publiques par les cabinets de conseil McKinsey,

vis-à-vis des géants de la finance, de leurs influenceurs et lobbyistes

déroulé le tapis rouge à cette entreprise. Qui a poussé la régulation des géants du numérique, monsieur le sénateur ? C'est la France ! Qui a convaincu le monde de mettre en place une fiscalité pour les géants du numérique, sous l'impulsion

Monsieur le président, mes chers collègues, je vais tenter par cette question de sortir du pessimisme ambiant ... Certes, la situation internationale est difficile, et les conséquences sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français sont notables. Les deux projets de loi que nous allons examiner ces prochains jours sont des réponses concrètes et immédiates aux défis que nous devrons surmonter. Pour autant, si les nuages sont bien là, ils ne recouvrent pas totalement notre ciel, bien au contraire ! Il y a de bonnes nouvelles, il faut aussi le dire, sur le front de l'emploi de l'apprentissage, mais aussi dans notre industrie. Pour la troisième année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Nous creusons même l'écart avec nos rivaux historiques, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Concrètement, cela veut dire que notre industrie a un avenir un avenir international, technologique, écologique et numérique, ce qui offre une bouffée d'air à nos emplois. La cinquième édition du sommet ne fait que confirmer cette reconquête industrielle. C'est ainsi que quatorze entreprises se sont engagées pour un montant global de 6,7 milliards d'euros et la création de 4 000 emplois

pour la fabrication de composants électroniques. Bref, c'est un investissement inédit pour notre industrie. La reconquête industrielle doit en effet être une priorité de ce gouvernement pour renforcer notre souveraineté économique. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire, les défaillances de nos chaînes de production à des pénuries de produits essentiels comme les médicaments, les masques ou les respirateurs. Nous avons bien vu qu'il était urgent de relocaliser un certain nombre de chaînes de valeur. Ces faiblesses doivent être derrière nous. Avec l'innovation, la régulation et la décarbonation, nous pouvons continuer à transformer notre industrie. Pour ce faire, nous comptons sur votre détermination et votre compétence, monsieur le ministre. Pourriez-vous nous décrire votre feuille de route pour faire de l'industrie un nouvel eldorado économique ?

dernières années ont conduit à un déclin industriel qu'on pensait inéluctable, et que les cinq dernières années ont permis d'enrayer. Je salue à cet ma prédécesseure, Mme Agnès Pannier-Runacher, qui a contribué, avec le Président de la République, avec le ministre de l'économie et des finances, mais surtout avec les industriels de tous les territoires, à enrayer le déclin industriel français, qui n'est pas une fatalité. Oui, le sommet a été un succès.

vous n'avez pas voulu augmenter les revenus du travail de manière significative pour les classes populaires et les classes moyennes. Plusieurs fois, mon groupe a regretté sur ces travées des mesures prises sans cohérence, toujours trop tard, toujours sous la contrainte, toujours le dos au mur. Plusieurs fois, sur ces travées, nous vous avons demandé un rééquilibrage de la fiscalité entre le travail et le capital, alors que vous l'avez sciemment déstabilisée par un hyperbouclier fiscal que même Nicolas Sarkozy, votre nouvel ami politique, n'aurait osé imaginer. au moins un sujet sur lequel on peut vous reconnaître une forme de constance, tant votre politique sur ce point a toujours favorisé les mêmes, par un miracle physique : le ruissellement vers le haut, vers les plus aisés Aujourd'hui, vous entamez un nouveau quinquennat, marqué par une situation économique inquiétante. Le mécanisme de revalorisation automatique du SMIC n'est plus suffisant pour compenser l'inflation. C'est le moment de changer de méthode renoncez à cette politique de fuite en avant, celle des chèques qui n'ouvrent aucun droit, à laquelle personne ne comprend plus rien ! Vous vous présentez comme un gouvernement qui est dans l'action et non dans l'incantation. Je vous le dis, madame la Première ministre : les Français demandent non pas l'aumône, mais une juste reconnaissance de leur travail. Pour répondre à cette attente, je vous soumets de nouveau deux solutions justes et efficaces : la revalorisation du SMIC à 1 500 euros et une grande conférence sociale pour augmenter les salaires. Pouvez-vous, madame Borne, expliquer clairement aux Français pourquoi vous vous opposez à ces deux propositions ?

la première priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat. Ce doit être aussi notre priorité commune. Depuis le premier jour, mon gouvernement est à l'action, dans la continuité de ce qui avait été fait par mon prédécesseur Jean Castex depuis l'automne dernier, sous l'autorité du Président de la République. Nous avons agi pour le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle que nous avons mis en place à l'automne dernier un bouclier tarifaire

L'action que nous avons menée, c'est aussi la remise sur les carburants. Sans cette remise, le prix d'un plein de 50 litres serait plus cher de 10 euros. Et nous avons agi avec l'indemnité inflation, avec la revalorisation du barème de l'indemnité kilométrique, avec une aide exceptionnelle sur le chèque énergie, autant de mesures qui ont protégé les Français, notamment les plus modestes et ceux qui travaillent. Monsieur le président Kanner,

pour l'ensemble des Français. La guerre en Ukraine dure, les perspectives économiques s'assombrissent, les prix continuent à monter. Nous voulons donc prendre de nouvelles mesures pour les protéger. C'est tout le sens des textes sur le pouvoir d'achat

d'augmenter les revenus du travail et de mieux partager la valeur, par exemple avec une baisse de charges pour les indépendants ou un triplement du plafond de la prime de pouvoir d'achat. Ils visent aussi à revaloriser les retraites les prestations sociales, et à aider les travailleurs pour lesquels la voiture est une nécessité. Et sur les salaires ? Bref, nous voulons agir globalement pour l'ensemble des Français. Je vous ai présenté nos propositions ; nous voulons en débattre avec le Parlement, mais nous serons attachés dans les discussions à venir à ce que ces propositions soient efficaces, c'est-à-dire qu'elles se traduisent par un impact rapide pour les Français, mais aussi responsables,

pour vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Au cours du mois de juin, dix jours de grêle ont ravagé 30 000 hectares de vignes sur l'ensemble des terroirs français,

Nous ne savons plus comment faire face à l'accumulation des difficultés. La crise diplomatique avec les États-Unis, la crise covid, avec la fermeture des bars et des restaurants, la crise climatique, la crise inflationniste : face à ces innombrables défis, les viticulteurs ont besoin d'un soutien massif du Gouvernement. J'ai une pensée également pour nos sylviculteurs, nos élus et pompiers girondins, qui se battent depuis hier soir sur le front de trois incendies dévastateurs. Je remercie M. le ministre Darmanin d'avoir décidé de s'y rendre tout à l'heure. À court terme, il semble inévitable de mettre en place un fonds d'urgence pour venir en aide non seulement aux viticulteurs, mais aussi, plus largement, aux agriculteurs, dont la trésorerie a disparu avec cette succession de crises. Nombre d'agriculteurs ont souscrit un prêt garanti par l'État (PGE), mais la situation actuelle transforme son remboursement en véritable couperet. Aussi, l'allongement généralisé des délais de remboursement des PGE est la seule solution

si le mode de calcul des références de production historique, fondé sur la moyenne olympique, ... Votre question ! ... ne permettent pas de tenir compte de l'enchaînement des aléas ayant frappé nos terres ces dernières années. Monsieur le ministre, quelles annonces pouvez-vous faire ici aujourd'hui pour prévenir les drames familiaux et entrepreneuriaux à venir ? La

à des médecins peu soucieux d'y défendre un service public universel de qualité ». Votre traitement d'urgence fait de nouveau la part belle au libéral en multipliant les différences de rémunération entre ceux qui exercent et restent à l'hôpital, assurant quasiment seuls la pénibilité de la permanence des soins, et ceux à qui vous n'imposez aucune obligation de prendre enfin leur part, tout en leur octroyant des surrémunérations horaires, creuse le différentiel, dégrade l'attractivité de l'hôpital et alimente le cycle des démissions et vacances de postes. Votre diagnostic est incomplet : il omet l'absence de lits d'hospitalisation, par exemple aux urgences pédopsychiatriques hospitaliser les enfants en détresse psychologique. En effet, vous continuez à fermer des lits ! Votre préconisation principale porte sur le tri des patients à l'entrée des urgences, alors que les SAMU sont déjà débordés et que 10 % des postes d'assistants de régulation médicale sont vacants. En Seine-Saint-Denis, depuis que l'on encourage à appeler le 15, seuls 8 % des appels peuvent être décrochés dans la minute.

s'inscrivent-elles dans votre vision des urgences, réduite aux seules urgences vitales- cela n'est pas notre conception -, ou bien, une fois l'été de tous les dangers passé, allez-vous enfin consentir à nous présenter un budget à la hauteur des besoins de santé des populations et des territoires ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Poncet Monge, ma mission, en tant que ministre de la santé, c'est de permettre à chaque Français d'être pris en charge de manière adéquate lorsque cela est nécessaire. Cette mission ne se limite pas, bien entendu, à l'urgence vitale, vous l'aurez compris. Je veux tout d'abord couper court à ce que j'entends parfois. Chaque Français continuera bien à être pris en charge dans le cadre de l'urgence et des soins non programmés là où ce sera le plus utile pour lui.

le parcours de soins le plus adapté. J'ai l'habitude de le dire : quand on a mal au genou depuis trois semaines, il vaut mieux aller voir son médecin traitant ou un médecin généraliste proche plutôt que d'aller dans un service d'urgence. Nos services d'urgence font face à une tension qui n'est pas seulement liée à leurs difficultés ou aux difficultés de l'hôpital. Il y a bien un enjeu systémique global d'organisation de l'offre de soins.

Je ne reviendrai pas sur les 41 mesures. Vous en proposez, madame la sénatrice, une 42, qui est de rouvrir des lits. Je vous rejoins totalement, mais, pour ouvrir des lits, il faut des soignants ; pour avoir des soignants, il faut qu'ils reviennent à l'hôpital ; pour qu'ils reviennent à l'hôpital, il faut qu'ils retrouvent du sens à leur métier. C'est là un objectif important. J'ai signé dimanche

sur deux éléments principaux. Pour la première fois, on reconnaît la notion de pénibilité, en particulier la pénibilité du travail de nuit. C'est une porte ouverte. Bien entendu, il faut aller plus loin. En ce qui concerne la permanence des soins, il ne vous aura pas échappé

Vous l'aurez compris, ma volonté est de faire travailler tout le monde ensemble : les soignants, les soignés, les élus, le privé et le public, en s'affranchissant des silos qui existent à ce

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. Monsieur le ministre des outre-mer, après plus de deux semaines de mobilisation et de négociation dans le cadre de la nouvelle convention « canne les planteurs réunionnais ont enfin obtenu gain de cause hier soir. Je vous remercie d'avoir pesé de tout votre poids pour que cette négociation aboutisse. C'est la fin d'un conflit qui aura duré longtemps, bien trop longtemps, comme c'est le cas malheureusement à chaque renégociation de cette convention depuis plus de vingt ans. Si agriculteurs et usiniers ont trouvé un accord global sur les six prochaines années, il n'en demeure pas moins que les acteurs de la filière restent très inquiets pour l'avenir de leur profession. leur profession. Ils n'ont pas obtenu satisfaction sur plusieurs points, notamment sur le fait que l'industriel Tereos refuse toujours d'adopter à La Réunion le même modèle coopératif qu'il applique en métropole, lequel garantit une meilleure répartition des richesses. Les planteurs regrettent également que l'État ne les accompagne pas davantage, au moins le temps que durera la situation actuelle, pour faire face aux prix des intrants, l'engrais notamment, qui ont été multipliés par trois ces derniers mois. Enfin, ils réclament toujours que la prime toujours que la prime bagasse soit revalorisée. Cette prime, actuellement de 14,50 euros par tonne de canne, n'a en effet pas évolué depuis 2015, alors que, pour des énergies polluantes telles que le charbon, le montant est passé de 80 euros à 400 euros. Au regard de ces inquiétudes légitimes et des enjeux cruciaux qui en découlent, monsieur le ministre, quelles actions pérennes comptez-vous mettre en oeuvre pour sauvegarder cette filière « canne », qui demeure plus que jamais au coeur d'une économie circulaire employant dans nos territoires ultramarins des milliers de nos concitoyens ?

Tout le monde a fait des efforts significatifs : Albioma pour revaloriser la prime bagasse- 3 euros de plus pour les planteurs -, les planteurs et Tereos pour aboutir à une répartition équilibrée des bénéfices- nous sommes allés chercher les bénéfices accumulés par Tereos pour les remettre dans la convention et pour répartir les bénéfices à l'avenir si bénéfices il y a. Dans le même temps, l'État a augmenté l'aide aux planteurs de 14 millions d'euros et confirmé l'aide à l'industriel de 28 millions d'euros. Le résultat est sans commune mesure avec ce qui préexistait, puisque, pour la première fois, le prix d'achat de la canne pourra être

Sur la signature particulière de Tereos à La Réunion, je répète ce que j'ai dit hier à l'Assemblée nationale : je travaillerai avec les autres ministres concernés à renforcer la transparence

Le ministère des outre-mer et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire vont désormais travailler sur la souveraineté alimentaire à travers la production animale et la production de fruits et légumes. Les premières discussions que j'ai eues avec le ministre chargé des comptes publics,

où j'ai souhaité rencontrer les équipes de la maternité pour voir comment se préparait l'été. Il s'agit d'un établissement de niveau 3, qui réalise plus de 4 000 accouchements par an, et qui prend en charge, notamment, des grossesses à risque. Je pense aux femmes atteintes de drépanocytose. Le constat que nous y avons fait est accablant.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la présidente Deroche, vous avez raison, le problème de notre système de santé est systémique. Au-delà de la crise conjoncturelle que nous vivons actuellement, c'est bien sur l'ensemble du système de santé qu'il faut faire peser nos efforts. Notre pays connaît depuis plusieurs années une réorganisation continue des maternités, sous l'effet, déjà, de contraintes de démographie médicale, mais aussi, et surtout, pour tenir compte d'exigences de sécurité et de qualité des soins que nous devons à l'ensemble de nos concitoyennes. Des inégalités persistent. Je vais lutter contre celles-ci, comme d'ailleurs, de façon générale, contre toutes les inégalités d'accès à la santé. En réponse à ces constats, nous agissons déjà pour mieux prendre en charge les femmes dans nos maternités, avec le déploiement en cours de maisons de naissance maisons de naissance expérimentales en voie de pérennisation pour une cible de vingt à court terme. Le projet d'extension des missions des centres périnataux de proximité vise à apporter une réponse au plus près des territoires. actions dans le champ de la santé de la femme et de l'enfant. Il y a également l'expérimentation d'équipes mobiles de néonatalogie à domicile, la mise en place pour les femmes issues de territoires isolés de la prise en charge d'un hébergement de proximité à la maternité, ainsi que des frais de transport. Nous renforçons aussi l'attractivité des métiers du soin, notamment pour les maternités. Je pense en particulier à la question de l'exercice mixte ville-hôpital pour les sages-femmes. Vous parlez de faire revenir des sages-femmes à l'hôpital. Les sages-femmes avec qui j'ai discuté quittent l'hôpital aussi à cause de la pénibilité de la permanence des soins. Je le répète, cette pénibilité de la permanence des soins ne doit pas porter seulement sur l'hôpital public ; elle doit être partagée entre le public et le privé. Les professionnels exerçant en maternité ont par ailleurs bénéficié de 12 millions d'euros de revalorisation « Ségur Les sages-femmes ont connu également une revalorisation complémentaire, portant la hausse de revenus à 500 euros par mois en moyenne. Nous poursuivons en outre des actions pour développer nos capacités de formation dans ces métiers et ces spécialités par l'ouverture de places,

et Républicain. Il y a six mois, le président Macron, devant le Parlement européen, a émis le souhait d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous avons été nombreux et nombreuses à applaudir à ce moment-là. Depuis lors, il y a eu l'effroyable décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a été pour nous un choc brutal. Aucune démocratie n'est désormais à l'abri : le lobby international anti-IVG, anti-choix, est puissant, il dispose de moyens financiers importants, de relais idéologiques, politiques et religieux. Personne ne peut dire ce qui se passera en France demain ou après-demain.

inscrire à l'ordre du jour un projet de loi constitutionnelle pour définitivement garantir dans la Constitution le droit à l'avortement et à la contraception

l'Histoire fourmille d'exemples de libertés fondamentales que l'on croyait acquises et qui ont été balayées comme des fétus de paille. Le cas américain nous rappelle que, même dans les grandes démocraties, ce que l'on croyait acquis depuis cinquante ans ne l'est pas Le droit à l'IVG est un droit fondamental, bien sûr, et personne- je dis bien : personne -ne peut envisager de retirer aux femmes le droit de disposer de leur corps.

Le droit à l'IVG est ici mieux protégé, et je sais que ma collègue Isabelle Rome se bat au quotidien pour donner à toutes les femmes un égal accès à celle-ci, mais, de grâce, ne prenons pas de C'est pourquoi, en tant que garde des sceaux, je soutiendrai avec force ces initiatives pour les voir aboutir. Le Parlement est dans son rôle ; le Gouvernement sera dans le sien pour qu'enfin le droit à l'IVG devienne un droit inaliénable.

sur l'accès à l'IVG. C'est la seule solution pour que vos engagements se concrétisent, pour que votre mandat à Matignon soit non pas simplement le mandat d'une deuxième femme Première ministre, mais le mandat d'une deuxième femme Première ministre qui a fait avancer les droits des femmes. Je vous le redemande : faites un projet de loi

Républicains. Ma question s'adresse à Mme la Première ministre, dans le prolongement de la question posée par ma collègue François Gatel. Madame la Première ministre, vous avez à plusieurs reprises, et notamment dans cette enceinte, mercredi dernier, lors de votre discours de politique générale, affirmé votre respect pour le Sénat et votre volonté de vous inspirer à l'avenir de ses travaux. En voici une occasion, à travers un sujet majeur qui préoccupe aujourd'hui les maires, à savoir l'objectif de zéro artificialisation nette, que l'on va donc appeler ZAN. Après avoir fait une trentaine de déplacements dans le pays, je peux vous dire que les élus sont en ébullition sur ce sujet.

tout le monde, puisqu'il n'y a aucune ingénierie mise à la disposition de nos élus pour atteindre cet objectif. Enfin, ils reprochent au pouvoir réglementaire, que vous incarnez, de revenir sur la loi. C'est quand même assez grave, quand on pense à la hiérarchie des normes- on peut encore prononcer ces mots

il me semblait que le début de réponse que j'avais fait à Mme Gatel permettait de vous donner une idée de notre détermination. Je vais donc aller un chouïa plus loin.

Sophie Primas, a communiqué le 6 juillet sur le retour des 1 242 questionnaires envoyés pour comprendre ce que les élus locaux reprochaient à ce début d'exécution du zéro artificialisation nette.

traiter les disparités territoriales, et avec quels moyens d'accompagnement financier. Votre première préconisation sur la pérennisation du fonds friches inscrite dans le plan de relance a d'ores et déjà fait l'objet d'un arbitrage favorable de la part de la Première ministre. À

sur lesquelles on peut travailler ! Alors, au-delà de la séance d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour que nous puissions avancer : la volonté est réelle, le cap donné par la Première ministre est clair et l'ambition est partagée Dont acte, monsieur le ministre, sachant que les élus locaux ont jusqu'au 22 octobre pour faire des propositions à leurs régions respectives. Il y a donc véritablement plus qu'urgence.

a été marquée par des événements d'une particulière gravité. Si le pire a pu être évité, les dysfonctionnements constatés ce jour-là ne doivent et ne peuvent pas être minimisés. Nous devons des explications à ceux qui en ont été victimes- je pense en particulier aux supporters du club de Liverpool -, mais aussi à ceux qui, depuis lors, s'interrogent sur la capacité de notre pays à organiser de grands événements sportifs, notamment la coupe du monde de rugby l'année prochaine et les jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Le Sénat, à travers ses commissions des lois et de la culture, de l'éducation et de la communication,

y faisions. Notre objectif était d'identifier de manière précise les dysfonctionnements, d'établir les responsabilités des uns et des autres et de faire des propositions pour éviter que cette situation ne se reproduise. Madame la Première ministre, votre parole a été rare sur ce sujet.

pour la réplique. Madame la Première ministre, monsieur le ministre, nous partageons votre souci de faire en sorte que les jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent dans les meilleures conditions possible.

205 délégations étrangères et 10 000 athlètes, à quoi s'ajoute la présence de nombreux chefs d'État, et tout cela devant 600 000 spectateurs. Les interrogations s'accumulent, enfin, sur la manière dont la Ville de Paris gère ces jeux. À ce jour, pas moins de 5 000 chantiers gangrènent la capitale. De nombreux élus parisiens réclament davantage de transparence dans la gestion de ce dossier, sans réponse de la maire de Paris. Même l'ancien ministre et champion olympique Guy Drut nous alerte sur les risques d'explosion des coûts et le manque de concertation.

Aussi, pouvez-vous, madame la Première ministre, confirmer que le Gouvernement a pris la pleine mesure de ce dossier et qu'il veille à « sécuriser le cadre budgétaire et financier des jeux », comme l'a réclamé la Cour des comptes ? La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur

vous l'avez dit, Paris 2024, c'est la promesse d'une grande fête, mais aussi un défi majeur : la livraison de l'ensemble de ces infrastructures.

lors, il serait de mauvaise manière de se défausser sur le Gouvernement, en considérant que la crise des finances locales viendrait justifier d'une manière ou d'une autre un appel à un coup de main particulier de notre part.

la fierté d'organiser ces jeux et le fait de revendiquer un certain nombre de décisions qui relèvent de la mairie ne doivent pas conduire à se défausser sur le Gouvernement de décisions qui sont prises à un autre échelon que le nôtre. La parole est à M. Pierre Charon, pour la réplique. Monsieur le ministre, vous êtes trop subtil pour ne pas avoir compris ma question Il ne s'agissait pas de me défausser ; je parlais surtout, bien évidemment, de la mauvaise gestion de la maire de Paris. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

a suscité une véritable déflagration dans le monde des Ehpad. Face aux manquements du groupe Orpea dans le soin porté aux résidents, face aux atteintes aux droits des salariés, face à la faiblesse documentée de l'action publique dans la surveillance de ces activités, le Sénat a mis en place une mission d'information sur le contrôle des Ehpad dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête.

Alors, monsieur le ministre de l'autonomie, ma question est simple et appelle une réponse tout aussi simple : le Gouvernement va-t-il prendre à bras-le-corps la question du grand âge et de la perte d'autonomie ? Va-t-il nous proposer un projet de loi

de ces sujets reposent sur les compétences des collectivités locales dont vous êtes les représentants. J'aurai aussi à coeur d'entretenir un dialogue permanent, transparent et de qualité avec les collectivités. vous l'avez dit, les urgences sont nombreuses dans ce secteur. Je connais parfaitement les attentes des personnes accompagnées, des familles, mais aussi des professionnels, dont je tiens à saluer l'engagement constant, particulièrement dans cette période difficile. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai

Entendez l'urgence des professionnels, qui la proclament depuis fort longtemps ! Entendez aussi l'urgence des familles, qui sont peut-être plus en demande encore depuis la crise sanitaire et qui ne peuvent pas attendre ! Le n'est plus possible, il nous faut un cadre de loi Monsieur le ministre, il y a quelques jours, dans mon département du Gard, le feu a consumé 900 hectares en près de vingt-quatre heures ! Bordezac, Bessèges, Gagnières, Générac ou encore Alès n'ont pas été épargnés. Aujourd'hui, de nombreux Gardois s'apprêtent à vivre leur été dans l'angoisse permanente de ces flammes. Je veux rendre ici un hommage appuyé aux sapeurs-pompiers mobilisés.

Monsieur le ministre, il faut absolument adapter nos textes à nos territoires. En effet, il arrive qu'au nom de la biodiversité des élus départementaux ou municipaux ne puissent débroussailler les abords des routes comme ils le souhaiteraient afin d'en faire de véritables coupe-feux. Il faut davantage laisser les préfets concilier ces deux objectifs qui, je tiens à le redire, ne sont pas antinomiques. Surtout, nos communes rurales du Gard s'étendent souvent sur de nombreux hectares ; elles ne peuvent assumer seules ce risque qui, malheureusement, est amené à s'amplifier. Le débroussaillement a un coût aussi important que son utilité, tout comme l'entretien des voies de défense de la Monsieur le ministre, vous conviendrez que les feux coïncident rarement avec les limites administratives ; la lutte contre les incendies doit donc pouvoir compter sur le soutien total de l'État.

Burgoa, comme vous, je voudrais rendre hommage aux services de l'État, aux sapeurs-pompiers, aux gendarmes et policiers, aux élus locaux, souvent des maires de communes rurales, qui, au risque de leur vie, préviennent les populations, organisent les secours et luttent des jours et des nuits contre ces feux,

Le 28 juin dernier, le Gouvernement a annoncé une revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Celle-ci est nécessaire afin de soutenir le pouvoir d'achat des agents. Toutefois, elle a un coût extrêmement lourd pour les collectivités territoriales : plus de 2 milliards d'euros par an. Cette hausse du point d'indice, décidée par l'État sans concertation et payée par les collectivités, intervient dans un contexte financier particulièrement difficile. À cette dépense de personnel s'ajoute l'explosion du coût de l'énergie et du carburant, des prix alimentaires ou de la construction. On entend également parler d'un désengagement de l'État sur les contrats aidés des parcours emploi compétences (PEC). Et ce n'est pas fini ! La semaine dernière, votre gouvernement a annoncé des entreprises (CVAE), soit 17 milliards d'euros en moins pour les collectivités. Pour rappel, le Président de la République veut leur imposer 10 milliards d'euros d'économie, alors même que le déficit de l'État, lui, ne cesse de se creuser depuis 2017

? Au-delà, quelles compensations comptez-vous mettre en place pour garantir aux collectivités leur capacité d'investissement et leur autonomie financière ?

locaux. Dans la continuité de vos propos, tous leurs représentants ont affirmé à quel point il était aujourd'hui nécessaire, après dix ans de gel du point d'indice, d'accorder une revalorisation à nos collaborateurs, dont nous vantons les mérites et pour lesquels il était nécessaire de faire un geste.

Mes chers collègues, sous réserve de la publication du décret portant modification du décret de convocation du Parlement en session extraordinaire et sous réserve de la publication de la lettre d'ordre du jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 21 juillet 2022, au matin, du projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Finlande